Chers collègues, la séance est ouverte. Compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, y a-t-il des observations sur son contenu. Il n'y en a pas. Il est donc adopté sous les réserves d'usage lors du jour. Appelle les réponses à des questions orales et la parole est d'abord au président Guillaume Gontard, qui a la parole pour 2 minutes. Ma question porte sur les pratiques douteuses du groupe avec dirigé par Monsieur Bernard Bensaïd. Réunissant 400 établissements et 12.000 salariés, notamment dans la santé, le médico-social. Ce groupe risque la faillite suite aux agissements de son patron. Pendant des années avec a connu une croissance effrénée et selon un ancien cadre du groupe. Monsieur Bernard Ahmed Saïd et comme un gamin qui joue au Monopoly cherchant à bâtir un empire qui deviendrait too Big to fail un empire étroitement contrôlée par Monsieur Bensaïd et ses proches. Le conseil d'administration est exclusivement composée des membres de sa famille et des salariés sous son influence. Pour faire grossir son groupe Monsieur Bensaïd va avoir l'habitude de vider la trésorerie des établissements qu'ils contrôlent la clinique mutualiste de Grenoble a qui en 2020 on a fait les frais. Le groupe avec lui doit déjà 6, 5 millions d'euros et récupère chaque année 1% du chiffre d'affaires ce qui est illégal pour un explique toutes les dépenses sont. Des lignes téléphoniques sont coupées, les astreintes de médecins ne sont pas payées, le bloc opératoire a été privé d'électrocardiogramme pendant 15 jours, la santé des patients est en danger. Partout en France les mêmes pratiques se répète fournisseurs et employés ne sont pas payés loyers ne sont pas honorés. Ces retards de paiement mettent des centaines de personnes en difficulté les procédures judiciaires pour un pays et non respect. Des normes s'accumulent. Le 12 janvier, Monsieur Bensaïd a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics mais il contrôle son groupe indirectement en octobre, la Première ministre assuré qu'il n'y aurait aucune complaisance des pouvoirs publics vis-à-vis de ce groupe. Si la justice doit continuer son travail. L'État ne peut rester attentiste. Attentiste et à Grenoble et syndicats de la clinique demande la nomination d'un administrateur provisoire. Ma question est donc simple, le gouvernement compte-t-il accepté cette demande. Merci. Merci cher collègue. Madame la Ministre c'est à vous. Monsieur le président, monsieur sénateur la situation financière et les pratiques de gestion du groupe avec font actuellement l'objet d'un suivi rapproché de l'État et en particulier des services du ministère de la santé mais aussi du ministère des solidarités afin d'avoir la vision la plus claire possible de son organisation juridique sa situation financière, notamment suite aux retards de paiement de salaires sur certaines entités du groupe. Une expertise indépendante a notamment été lancé sur ce point avec contrôle en effet des établissements de santé, mais également de nombreux organismes privés titulaires d'autorisation d'exploitation de SMS, parmi lesquels des Ehpads, des résidences autonomie des Siad et des stades. S'il ne m'appartient pas de commenter l'enquête pénale en cours. Nous pouvons assurer que sur le plan administratif. Des actions sont en cours afin d'une part de garantir la continuité d'activité des établissements menacés et d'autre part de s'assurer de la sécurité et de la qualité des prises en charge à titre d'exemple, 13 des 18 et pas du groupe avec ont fait l'objet d'au moins un contrôle en 2022. D'autres concours de contrôles complémentaires sont programmés dans les mois à venir dans le cadre du plan national d'inspection de contrôle des 700.500 épate de francs sur deux ans. Engagé à la suite du déclenchement de l'affaire Orpea. Concernant les établissements sanitaires, les ARS bien informés des actions en cours priorisent la continuité des soins dans les établissements concernés. Par ailleurs, le gouvernement a d'ores et déjà engagé d'importantes mesures structurelles visant à la moralisation du secteur privé lucratif. À cette fin, l'article 62 de la FSS 2023 comporte un large panel de nouvelles mesures législatives en ce sens avec des obligations de transparence et de contrôle renforcé pour les établissements avec parallèlement un renforcement des capacités des autorités de contrôle faisant respecter ses obligations dans la continuité de ses premières actions. D'autres mesures importantes sont actuellement en préparation, visant notamment à préciser les changements importants de l'activité, l'organisation la direction où le flacon. Le fonctionnement des établissements médico-sociaux, mais aussi renforcer les sanctions pénales mentionné au code de l'action sociale et des familles en cas de manquement aux obligations fixées par ce dernier. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Président, vous avez eu une dizaine de secondes. Oui merci madame la ministre. J'entends ce ce suivi rapproché mais j'aurais bien voulu avoir une réponse et notamment allez vous déclenchez une inspection par l'IGAS et conclura à la nomination d'un administrateur provisoire s'est fait ailleurs et dans d'autres établissements et je pense que là il y a réellement urgence. Très bien. La parole est maintenant Jean-Luc Fichet, pour la seconde question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Lutter contre l'intérim médical abusif. C'est un des aspects de la loi Rist que nous soutenons totalement. Il faut stopper les abus indécent des mercenaires. Mais voilà, la loi s'arrête à mi-chemin et ne crée aucune obligation aux professionnels de santé qui ont ce type de pratique. Les intérimaires ont un coût de 3 millions d'euros pour le seul hôpital de Morlaix. 2000 à 5000 euros pour une garde de 24h. Ces tarifs sont une insulte aux médecins et spécialistes qui chaque jour se consacrent souvent dans des conditions difficiles à leurs patients pour un salaire bien moindre dans les mois à venir pèse la menace de voir les médecins intérimaires refusé l'missions qui leur était dévolu. On va en mesurer les conséquences avec par exemple la menace de la maternité de Morlaix faute de la présence d'anesthésistes pour maintenir la ligne de garde. La fermeture de 6 blocs opératoires ne fonctionnant qu'avec des intérimaires au CHU de Brest. Les syndicats nous alerte, madame la Ministre, il n'y a aucune anticipation de la part du gouvernement alors qu'une loi existe depuis 2017, loi jamais appliquée. Le ministre-Brown a déclaré hier au Sénat qu'aucun territoire ne serait laissé sans solution. Si la situation se détériorer. La situation se dégrade. Quelles mesures le gouvernement entend-il donc mettre en place en urgence pour éviter la possible fermeture de services hospitaliers comme à Morlaix ou Brest. Ne pensez-vous pas Madame la Ministre qu'il est urgent de créer des obligations à des professionnels pour qui l'argent passe avant le besoin vital des patients et dont les études sont totalement financées par de l'argent. Public. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, les dérives de l'intérêt médical représente un poids financier important pour l'hôpital public avec certaines rémunérations de l'Ordre de 3000 euros pour 24h. Ces situations engendrent également une iniquité vis-à-vis des praticiens qui s'investissent durablement à l'hôpital ainsi l'intérêt médical fait l'objet d'un plafonnement depuis la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 à un montant de 1170 euros brut pour 24h. Cependant les infractions à cette réglementation n'ont cessé de se développer ces dernières années. Ainsi la loi Rist du 26 avril 2021 que vous avez cité vise à rétablir un équilibre et une équité en faisant respecter ce cadre réglementaire, je le rappelle, notre politique n'est pas de lutter contre l'intérim qui peut parfois représenter une solution à certaines situations de tension conjoncturelle aux ressources humaines mais contre ces dérives aussi l'application des dispositions de la loi prévue à partir du 3 avril prochain font l'objet de travaux préparatoires importants et donc d'anticipation Monsieur le sénateur, contrairement à ce que vous avez dit les services du ministère de la Santé et des ARS travaillent en étroite liaison avec les établissements publics et le réseau des finances publiques pour préparer l'entrée en vigueur des contrôles et anticiper les conséquences sur l'offre de soins localement. élus locaux et par les élus locaux et parlementaires soit. Dans le cadre de ce travail des diagnostics territoriaux ont été établis pour identifier au cas par cas les problèmes éventuels et des solutions adaptées au maintien de la continuité des soins. Des concertations sur le secteur privé sont par ailleurs en cours pour définir des modes de fonctionnement solidaire enfin les dispositif indemnitaire et plus largement de rémunération ont été créés pour renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier les statuts des praticiens hospitaliers et contractuels ont été revalorisés des indemnités spécifiques ont été très créé telles que la prime de solidarité territoriale et les mesures de majoration des indemnités de garde mise en place à l'été, ont été prolongées cet hiver. Merci, madame la Ministre, Monsieur Fischer. parce que ceux-ci ne veulent plus venir, faute d'être grassement payés et donc on va se retrouver avec des services qui vont fermer et la question c'est, que pensez-vous faire pour que ses services ne ferme pas et pour que les hôpitaux fonctionnent dans des conditions correctes au bénéfice de l'ensemble des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Maintenant, la parole est à monsieur Patrice Joly. Merci monsieur le président, madame la ministre, je me permets de vous alerter sur les conséquences dramatiques de la suspension décidée depuis décembre dernier de la maternité d'autant l'application stricte des décrets de 1998 qui prévoit la fermeture des maternités enregistrant moins de 300 accouchements par an à multiplier par 2 le nombre de futures mères résidant à plus de 45 minutes d'une maternité, or un trajet de plus de 45 minutes

désormais à plus de 45 minutes d'une maternité pour certaines d'entre elles d'ailleurs la durée dépasse aujourd'hui 1h15 dans ces conditions les habitants. Habitants et élus, nous nous élevons contre telle décision qui ajoute encore plus à la désertification médicale déjà existants, alors même que la Cour des comptes avait précisé en 2014 que le seuil de 300 accouchements n'avait fait l'objet d'aucune étude spécifique lors de sa fixation de plus la solution proposée par par l'AS de création d'un centre de périnatalité a autant y à Château-Chinon soulève de sérieux doutes sur 3 points sur la paie sa pérennité au regard de l'expérience malheureuse de sur Loire ou après la fermeture de la maternité en 2018, le CCP qui lui a succédé est aujourd'hui fermé depuis 2 ans sur le caractère dégradé de la réponse puisque un centre se limite à assurer le suivi gynécologique et obstétrique sur l'insécurité, liée au délai d'accès la maternité conçu un enjeu. Majeur pardon Madame Dominique unique moyen de garantir aux futures mères une prise en charge descendent de leurs accouchements et de maintenir sur ce territoire la maternité. Autant je vous remercie. Merci la parole est à la manie madame la Ministre. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur d'abord excusez François Braun, qui ne peut être présent, il m'a pas prié de vous fournir les éléments suivants, la situation de la maternité d'autant fait l'objet d'un suivi rapproché tant au niveau du ministère de la Santé que localement au cours des derniers mois qui ont précédé la fermeture qui je le rappelle est temporaire de cette maternité. L'engagement de l'ARS, Bourgogne, Franche-Comté, ainsi que celui des autres acteurs du territoire a été constant pour tenter d'identifier des leviers de réponse aux problème de personnel tout en insécurité tout en assurant la sécurité des femmes enceintes et des nouveau-nés la persistance de graves défauts de continuité médicale au sein de l'établissement conjuguées aux problèmes de sécurité que ceci était susceptible d'engendrer ont toutefois conduit l'ARS mi-décembre dernier à une première décision de fermeture temporaire de la structure qui a été reconduite mi-janvier. Encore une fois dans le seul but de garantir la sécurité des parturientes et des nouveaux-nés. Dans ce contexte de démographie des professionnels de santé en graves tensions l'ARS concentre tous ses efforts afin de ne laisser aucun territoire du Morvan sans solution. Il s'agit désormais, dans le cadre d'une réflexion intégrant toutes les parties prenantes concernées ARS soignants, élus de construire des réponses adaptées aux besoins de santé de la population, prenant en compte la situation particulière du Territoire particulièrement enclavé afin de laisser tout le temps nécessaire à ce travail local avant qu'il ne soit définitivement statuer sur l'avenir de la peine maternité le ministre François Braun a annoncé mi-février. Le report de la suspension définitive de la maternité d'Autun et la réouverture d'une concertation locale sur l'avenir de l'établissement. La réflexion porte actuellement sur la formalisation d'un accord partenarial pour la création d'une maternité territoriale Nièvre et Saône-et-Loire visant à offrir une réponse sécurisée et coordonnée pour les parturientes et leur nouveau-né, il est essentiel et nous y serons extrêmement attentifs que les femmes résidant sur ce territoire bénéficie d'une solution satisfaisante à leur grossesse plusieurs solutions telles que la création d'un SMUR obstétrical sont actuellement étudiées en ce sens en appui à ces réflexions local. Tout est mis en oeuvre à l'échelle nationale pour qu'une fermeture de maternité ne se traduisent pas par une importante perte d'emploi ou par de moins bonnes conditions de suivi pour les femmes et leurs nouveaux-nés avec des solutions construites autour de centre périnatal de proximité rénovés et attractifs et d'hébergement des femmes en proximité des maternités référente.

répondre aux exigences votre proposez vos propositions formulées par le corps médical experts maternité ou si on veut assurer la sécurité sanitaire des territoires ruraux et du Morvan, en particulier je m'apprête à déposer une PPL tendant à garantir un droit nette dans tous les territoires. Je vous remercie. Très bien. La parole est maintenant la présidente Catherine Deroche. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame le ministre et porte sur le. La gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux, autrement dit les Dasri. Constatant les pratiques de tri de ces déchets qui sont très hétérogènes. La direction générale de la Santé a légitimement en décidé d'entamer la révision du Guide 2009 sur la gestion de ces déchets pour les professionnels de santé et cette révision est plus que nécessaire aujourd'hui puisque cette filière constitue en effet un maillon important dans notre chaîne de soins, alors si la simplification des pratiques de très impératif. Celle-ci doit néanmoins se faire en garantissant la protection des de la santé des agents qui sont au contact de ces déchets. Temps durant le transport que à l'occasion de leur élimination. Cependant, il semblerait que la DGS envisage. D'orienter les déchets à risques infectieux vers la file hier des ordures ménagères, ce qui n'est pas sans risque et et les agents en charge de collecter, traiter les ordures ménagères ne bénéficient pas en effet forcément de protection individuelle équivalente à leurs homologues de la filière Dasri et peuvent être exposés en effet à des coupures à des objets ont de sang. Par ailleurs, il y a, c'est également un risque environnemental puisque les camions des ordures ménagères ne sont pas habilités à transporter des matières dangereuses que pas le cas tous les Dasri mais ça peut l'être au regard de leur absence d'étanchéité. Sans compter des horreurs de tri nouvelle qui pourrait naître. Donc je voulais savoir. Ce que le gouvernement pense de cette. Solution que préconise la DGS d'orienter vers les ordures ménagères. Merci madame la ministre, votre réponse. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Le guide de collecte et d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 10 Dasri nécessite une actualisation notamment des pratiques de tri qu'il recommande qui incite fortement à éliminer tout déchets de soins dans la filière des Dasri qu'ils soient ou non dangereux et ou infectieux aussi ces recommandations doivent être plus cohérente avec les objectifs environnementaux de la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire auxquelles doivent répondre les producteurs de déchets. Les pratiques de tri doivent également évoluer afin de répondre aux enjeux aux objectifs de l'action 14 du Ségur de la santé publique. Accélérer la transition écologique à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux qui vise à réduire le coût des déchets pour les établissements de santé. Les Dasri ayant un coût d'élimination en moyenne 2 fois supérieur au coût de l'émission des déchets d'activités des soins assimilés aux ordures ménagères dit down ainsi le ministère de la Santé a initié en juillet 2022, la révision de ce guide attendu par l'ensemble des secteurs. Un groupe de travail national piloté par la DGS et la DGOS a été constitué avec l'ensemble des parties prenantes de la filière dont les professionnels de la collecte et du traitement des déchets. La protection des travailleurs de la population et de l'environnement et le principe fondateur de la filière, la filière des Dasri et sera donc prioritaire dans le cadre des travaux menés une saisine du Haut Conseil de la santé publique sur ces questions est actuellement en cours, elle permettra de s'assurer que les conditions de mise en oeuvre des évolutions des pratiques de tri sont bien à même de garantir la sécurité sanitaire de la filière des Dasri comme celle de la filière des Dom. Les travaux du groupe de travail national prévoit également la mise à disposition d'outils pratiques d'aide au tri des déchets d'activités des soins à destination des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux ces travaux feront prochainement l'objet d'un point d'étape à l'occasion d'une réunion que je compte organiser en avril, elle sera consacrée aux différents chantiers relatifs à la transition écologique en santé. Merci madame la ministre. Et merci pour votre actualité dans la durée des réponses. Madame la présidente. Oui merci madame la ministre. On sera attentif, en effet je j'ai entendu tout ce que vous dites et je partage largement mais il faut être très très vigilant en effet sur la formation à la gestion des déchets aussi sur les risques que l'on a de modifier une pratique. Bien rodée, même si j'ai entendu les observations que vous faites. Quant à cette pratique. Donc nous attendons. C'est entendu, la parole est maintenant madame Annie Le Houerou pour sa question et pour 2 minutes. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre. La nouvelle carte scolaire des Côtes d'Armor prévoit la fermeture de 44 classes, 13% des communes du département sont concernés. Je ne peux tout de la cité pour Ivo la Roche dit et cetera. Ces annonces de fermetures font l'effet d'une déflagration au sein de la communauté éducative car elle porte atteinte à la promesse républicaine que représente l'école publique, les élus engagent la dynamique de revitalisation de leur commune grâce à des investissements importants et soutenu par l'État alors fermer une classe et tout simplement incompris par la population qui voit s'éteindre la lueur d'espoir cette attractivité par l'école est fondamentale car elle a un effet d'entraînement sur un panel de services médecin personnel soignant, entreprise, emploi local. La carte scolaire proposée fait fi des investissements qui ont été réalisés pour adapter les écoles à l'accueil d'élèves à particularité ou à la spécificité des classes maternelles ou élémentaires Saint-Brieuc à une fermeture, alors que les enfants handicapés accueillis ne sont pas comptabilisées des communes sont situées en zone de revitalisation rurale. Ah elle ne dispose pas d'accueil collectif de la petite enfance et accueille des enfants que vous ne comptait pas

par classes en élémentaire. Alors que la France est déjà à la traîne en Europe. En réalité, les moyens alloués ne sont pas à la hauteur des besoins et vous contraignent à une gestion arithmétique sans tenir compte des contextes locaux et de l'équilibre par niveau travailler en perspective avec la communauté éducative, les élus, des parents d'élèves sur un projet éducatif pluriannuel éviterait ces couperet annuel les mères vivent très mal cette situation. Ils sont prêts à rendre leur écharpe républicaine. Madame la ministre, je vous demande de réexaminer cette carte. Je vous demande un moratoire pour Les RPI ne reniait pas votre engagement de 20 22 élèves maxi par classe. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, le héros. Madame la sénatrice, après une baisse démographique de 300.000 élèves sur les 5 dernières années. 500.000 élèves de moins sont attendus d'ici à 2027, en raison de la priorité donnée à l'école par le gouvernement. Il fait donc le choix de préserver les moyens d'enseignement en faveur du redéploiement permettant déjà d'améliorer le taux d'encadrement du 1er degré mais également de stabiliser ceux du second degré et de poursuivre les politiques prioritaires dans le département des Côtes d'Armor et en dépit d'un contexte de baisse démographique des effets des élèves des effectifs élèves, soit 3148 élèves de moins depuis la rentrée 2017 les taux d'encadrement ont été. Ainsi, le nombre d'élèves par classe était de 21,20 à la rentrée 2022 à la rentrée 2023, les prévisions d'effectifs confirme cette baisse démographique avec 478 élèves de moins attendus dans les écoles du département. Cette baisse, elle concerne l'ensemble du territoire et plus particulièrement les circonscriptions de Lannion Lambel et Loudéac qui affiche des variations d'effectifs comprises entre moins 3,5 et moins de cinq. Certains secteurs sont très touchés par cette baisse démographique dans des écoles, y compris dans des regroupements pédagogiques intercommunaux pays dans lesquels les moyenne d'élèves par RPI reste faible, voire très faible. Après un examen attentif des derniers éléments apportés. Concernant la situation du RPI de très mail Lanvellec plus furent le directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor a suspendu la mesure de fermeture de classes pour la rentrée prochaine 2023. En outre, comme chaque année si le processus de préparation de rentrée commence en janvier. Il se poursuit jusqu'à la rentrée de septembre avec certaines situations qui pourront être revues en fonction des effectifs des élèves enfin je voudrais Madame la sénatrice vous dire que dans ce contexte de baisse démographique. Une réflexion est partagé sur l'école rurale de demain entre les élus et les différents services déconcentrés de l'État a été donc proposer. Réflexion à laquelle entre autres l'Association des maires de France a répondu favorablement, je vous remercie. dans l'école inclusive entrer en application le 1er septembre 2021. La grille indiciaire, des AESH est devenue obsolète en moins d'un an. Actuellement seuls 2 points d'indice sépare un AESH en CDI dans sa de 9ème année d'exercice d'un AESH en CDD dans sa première année d'exercice, alors qu'à l'entrée en vigueur de la grille, cet écart était de 20. Le tassement de la grille supprime par conséquent toute réévaluation et la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour ces personnels de plus leur temps de travail incomplet, le plus souvent imposé par des choix académique est synonyme de salaire incomplet et pour la grande majorité de SMIC incomplet. Par ailleurs, les dispositions de la circulaire du 5 juin 2019, définissant le cadre de gestion des AESH notamment celles relatives au calcul de la quotité de service ne sont toujours pas appliquées dans plusieurs académies dont celle de Besançon. Nombre d'AESH sont ainsi rémunérés pour une inférieure à celle correspondant à leur temps de travail effectif de la même manière les heures de fractionnement prévue à l'article 1er du décret du 26 octobre 84 ne leur sont pas accordé dans toutes les académies. Vous en conviendrez. Il n'est pas normal que les droits des AESH ne soit pas respecté. De la même façon sur tout notre territoire. Les inégalités de traitement d'une académie à l'autre, voire d'un département à l'autre doivent être corrigées au regard de ces éléments, je souhaiterais savoir quelles sont les intentions du gouvernement pour améliorer la situation professionnelle des AESH et mettre fin au NYSE et aux inégalités de traitement. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Jacques mais. Vous le savez, l'école inclusive est une priorité constante du ministère de l'éducation nationale et du gouvernement et la situation matérielle des AESH est un sujet majeur majeur d'attention. Je rappelle que 4000 postes d'AESH ont été créés au rentrée scolaire 2022 et 2023 et que les AESH ont bénéficié de la création d'une 10 d'une grille indiciaire. En septembre 2021 que vous évoquez, leur donnant une meilleure lisibilité et une amélioration de leur parcours professionnel, ce sont ainsi 150 millions d'euros qui ont été mobilisés pour l'amélioration de leur rémunération. Au cours de des 2 années 2021 et 2022, la loi de finances initiale pour 2023 a par ailleurs prévu une enveloppe de 80 millions d'euros pour revaloriser à hauteur de plus de 10% la rémunération de l'ensemble des AESH. Au 1er septembre 2023, soit plus de 240 millions d'euros en année pleine depuis le 1er janvier 2023 les AESH exerçant dans une école ou établissements relevant d'un réseau d'éducation prioritaire peuvent par ailleurs bénéficier d'une indemnité de suggestions annuel de Miss 106 euros les AESH exerçant elle en. Plus peuvent bénéficier d'une indemnité de suggestions de 3263 euros en parts fixe et d'eau, plus 448 euros par modulable. La loi dite Victor que votre assemblée a définitivement adopté le 16 décembre dernier permet par ailleurs aux AESH d'être recruté en CDI au bout de 3 années d'exercice dans des conditions qui seront prochainement précisées par décret la circulaire définissant le cadre de gestion des AESH du 5 juin 2019 que vous évoquez vise notamment à clarifier et harmoniser sur l'ensemble du territoire, les modalités de décompte de leur temps de travail afin d'assurer la reconnaissance de toutes les activités effectuées cette clarification associé à la prise en compte des activités connexes améliorant la rémunération des AESH est aussi fonction de la quantité de horaires travailler au-delà. L'objectif, vous le savez, c'est de proposer un contrat à temps de travail hebdomadaire de 35 heures pour celles et ceux qui le souhaitent, ce qui représentera un gain substantiel de revenus. Et un travail est prévue pour. Déterminer les missions qu'on mette l'inventaire avec des conclusions qui seront annoncées au printemps dans le cadre de la conférence nationale du handicap. Merci pour votre question. Merci madame la ministre, madame. Donc, chers collègues, vous avez quelques secondes si vous voulez souhaiter. Merci monsieur le président. Oui, je voulais vraiment insisté sur l'importance du travail qu'elles fournissent dans ces écoles et on voit bien que le regard sur les personnes en situation de handicap évolue et je pense qu'elles en font partie. merci de prendre en compte leurs demandes. Merci beaucoup. La parole maintenant à Madame Laure Darcos pour sa question. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée de l'enseignement et la formation professionnelle, madame la Ministre, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi l'Epide est un acteur reconnu dans le domaine de l'insertion des jeunes majeurs. Peu ou pas qualifiés et en voie de marginalisation. Plus de 3000 d'entre eux sont admis chaque année dans un des 20 centres, implantés en France dont celui de Brétigny-sur-Orge, dans mon département. Parmi ces volontaires motivés désireux de rompre avec la fatalité de l'échec, 30% sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. La prise en charge au sein de l'Epide et globale. Ils bénéficient d'un accompagnement sanitaire et sociale reçoivent un enseignement général, et spécialisé ainsi qu'une éducation à la citoyenneté et sont préparés pour l'emploi grâce à des périodes d'immersion dans le monde professionnel. L'importance attachée à la formation des volontaires à l'insertion est un atout pour les futurs employeurs les compétences acquises dans le cadre de leur parcours étant directement transférables dans les entreprises pour autant d'épiques pâtit d'une visibilité encore insuffisante. Parmi les dispositifs proposés aux jeunes sans qualification ni diplôme et auprès des opérateurs chargés de l'orientation de ces publics fragilisés dans ce contexte, je considère qu'il serait particulièrement judicieux de leur octroyer le statut de stagiaire de la formation professionnelle, dans bénéficie dont bénéficient les jeunes gens sous contrat de volontaires stagiaire du service militaire volontaire qui comme vous le savez, est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle très similaire à celui proposé au sein des centres Epide indéniablement, ce serait le gage d'une plus grande implication financière des régions auprès des jeunes et de l'Epide en tant qu'organisme disposant de la formation professionnelle. Entendez-vous Madame la Ministre mettre à l'étude cette proposition qui répond à une attente réelle des professionnels en charge de l'accompagnement de ces adultes en devenir et je vous invite quand vous le souhaitez à venir visiter mon centre à Brétigny. Je vous remercie de votre réponse. Madame le Ministre c'est à vous. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la la sénatrice Darcos. Les jeunes effectivement accueilli au sein de l'Epide ont le statut, vous l'avez dit de volontaires pour l'insertion et le volontaire le volontaire pour l'insertion perçoit une allocation qui a été valorisées afin d'être aligné sur le montant d'autres allocations d'insertion professionnelle. Les piles est un dispositif d'accompagnement qui organise des formations de remise à niveau scolaire et des actions d'insertion à destination de d'un public dont vous avez fort bien décrit et le profil qui souvent rencontrent des difficultés multiples notamment comportementale comportementale sociales qui sont sortis du système scolaire, qui sont souvent sans diplôme ni qualification et qui sont potentiellement en voie de marginalisation. L'encadrement de l'Epide, même s'il peut être inspirée du modèle militaire. Il s'en distingue par la mise en oeuvre d'une modalité de pédagogie originale qui souvent Ali suivi individuel dynamique du collectif mais aussi un accompagnement pluridisciplinaire pour accompagner toutes les difficultés que j'évoquais à l'instant les dispositions garantissent je crois un parcours de qualité pour ces jeunes accompagnés qui est souvent très personnalisé et si vous comparez ce dispositif au service militaire volontaire dont les volontaires dispose de la qualité de stagiaire de la formation professionnelle lors de leurs actions de formation en milieu civil. Qui font partie intégrante de leur parcours. C'est finalement à contrario de de l'Epide où le suivi d'une formation qualifiante ou diplômante constituerait une sortie positive finalement dont une sortie donc de l'Epide. C'est donc à ce seul moment que le jeune pourrait disposer de cette qualité de stagiaire de la formation professionnelle. La visibilité de l'Epide et je crois qu'elle s'est nettement améliorée et nous devons poursuit cette amélioration à ce titre, il y a différents chantiers qui ont été engagées en 2022, celui d'ouverture de l'ouverture des centres Epide le end permettant l'hébergement de jeunes, 7 jours sur 7 mais également de l'élargissement de l'accès aux dispositifs aux mineurs jeunes sans-domicile-fixe et bachelier éloignés de l'emploi. Et l'implication des équipes des centres et des et des ministères de tutelle ont aussi permis de faire grimper le taux d'occupation de l'des établissements à 91,1% au 31 décembre 2022 pour un total de 4291 volontaire pour l'insertion accueillis sur l'année, soit un record depuis la création des Epide et comme vous je le salue avec plaisir pour cette visite de votre épisode. Merci à très bientôt. Merci madame la ministre, qui, vous vous souvenez que le temps de réponse et de deux minutes et pas 2 minutes et demie. Madame. Madame Darcos. Non non mais je, je vous remercie pour votre réponse. Bon je je je j'aimerais bien en effet qu'on puisse. Creuser un peu plus cette, cette idée de statut. Exemple simple hein, ça leur permettrait même de bénéficier de tarifs réduits dans les transports, notamment l'Île-de-France, ils en pâtissent beaucoup ça n'est pas normal qu'il ne puisse pas avoir du coup le même statut que en effet les autres stagiaires de l'sa son professionnel. Entendu. La parole est maintenant monsieur Patrick Chaize pour sa question. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur le rapport du gouvernement au Parlement d'octobre 2022 et concernant la rémunération pour copie privée. Créée en 1985, la rémunération pour copie privée vise à compenser pour les ayants droit le préjudice lié à la copie de titre à titre privé de leurs Oeuvres. Une mission de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles à préparer le rapport du gouvernement au Parlement demandé dans le cadre de ma loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et remis celui-ci au Parlement en octobre 2022. Cette mission formule une série de propositions au nombres de 22 à plusieurs niveaux afin d'une part d'améliorer la gouvernance du dispositif en permettant une meilleure participation des parties prenantes et un enrichissement de la collégialité des décisions. D'autre part d'adapter le mode de calcul de la rémunération pour copie privée à la réalité des usages culturels et dans l'améliorer la transparence et l'acceptabilité et enfin de simplifier les exonérations et remboursement des usages professionnels de supports d'enregistrement. Si le dispositif rémunération pour copie privée présentent des marges d'amélioration, il apparaît en revanche fragilisé dans un contexte de transformation des usages introduite par le streaming et de développement d'utilisation des appareils reconditionnés suivant ces éléments et l'ambition de France station verte. Pouvez-vous m'indiquer les suites que vous entendez réservé au rapport du gouvernement au Parlement sur la révélation rémunération copie privée je vous remercie. Madame la Ministre, l'ancien rapporteur de la loi qui a créé cette rémunération vous écoute dans la réponse avec intérêt. Merci, monsieur le Président, j'entends la la haute pression que que vous mettez sur les épaules mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur chaises effectivement vous l'avez rappelé depuis 1985 la rémunération pour copie privée participe activement à la rémunération des ayants droit et au financement de de la vie culturelle. La loi du 15 novembre 2021 dont vous étiez, à l'initiative prévoit la transmission au Parlement d'un rapport portant sur ce sujet. Celui-ci a été réalisé par l'Inspection générale des affaires culturelles, ainsi que l'inspection générale des finances. Et a rendu public le 31 octobre dernier, ce rapport qui constate. Que le dispositif de rémunération pour copie privée présentent des marges d'amélioration. Il formule ainsi plusieurs recommandations, vous les avez rappelées, pour majoration. Pour la majorité, relève de la compétence de la commission dite copie privée. Le gouvernement se félicite de cette décision prise en janvier dernier par cette commission de travailler sur cette mise en oeuvre de ces recommandations. Cette dernière a ainsi mis à l'ordre du jour de sa prochaine séance en mars la modification du règlement son règlement intérieur et va également engager une réflexion sur les nouvelles améliorations à apporter dans son fonctionnement. En ce qui concerne l'adaptation du calcul de la rémunération à la réalité des usages. La Commission s'attachera principalement à refondre les Usa. Les études d'usage des principaux supports assujettis et a réagi à réexaminer les modalités de calcul de la rémunération. Le président de la commission devrait présenter lors de la prochaine réunion. Un document de cadrage. À cet effet pour un une meilleur usage. Téléphonique tablettes ainsi qu'un document de cadrage des valeurs de référence pour ce qui est des conditions d'exonération de certains supports destinés au marché au seul marché professionnel la Commission s'est engagée à à mener des discussions sur la possibilité d'exclure du Champ de la rémunération certains supports par nature destiné au seul marché professionnel et afin de garantir la réussite de ces chantiers. La ministre de la culture et le Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications ont fait droit à la demande du président de la commission tendant à ce que les 2 inspections ayant produit rapport soit désigné en appui du processus de mise en oeuvre de recommandations du rapport par la commission une la démission a été signé, donc le 22 février dernier. Obama dans le ministre de cette réponse, mais pour le dire aussi qu'il y a urgence effectivement pour faire en sorte que l'acceptabilité de cette redevance copie privée soit donc partager et que les effets sur notamment l'environnement dans le cadre des matériels reconditionné puissent aussi être efficace. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant madame Marie-Pierre Richer. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre je souhaite attirer votre attention sur les bénéficiaires des chèques énergie logeant en résidence pour personnes âgées dans la mesure où il existe une différence de traitement de ces chèques en fonction du statut juridique des établissements accueillant les personnes âgées. En effet, si cette disposition destinée à aider au paiement des factures d'énergie consacrés au logement est accordée à toutes les personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain montant son profit varie en fonction de leur mode de résidence. Si celles-ci occupent leur logement elle pour l'imputer sans difficulté sur le montant de la facture de leurs fournisseurs. En revanche, c'est en raison de leur âge, elle réside dans un établissement adapté à leur état de santé le bénéfice. Le bénéfice du chèque énergie qu'elles perçoivent varier en fonction de la nature des établissements, certains comme les EPHAD ou les résidences sociales sont autorisés en vertu de la loi à en bénéficier. Afin de diminuer le montant des factures de charges adressé aux résidents d'autres en revanche se voient refuser ce droit comme c'est le cas des résidences seniors ceci génère une inégalité de traitement au détriment de personnes généralement de situation modeste que rien ne justifie. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez m'informer des mesures que vous entendez prendre pour mettre fin à cette situation, je vous remercie. Madame la Ministre déléguée. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous, madame la sénatrice. Richard vous attirer l'attention du gouvernement sur la différence de traitement constaté s'agissant du chèque énergie en fonction du statut juridique des établissements accueillant des personnes âgées. Le chèque énergie comme vous. Savez bien et d'une aide de l'État attribuée aux ménages modestes pour les aider à payer les factures d'énergie leur logement ou leur travaux d'ailleurs de rénovation énergétique. Il a été généralisé en 2018 et il est effectivement attribués selon les revenus. La composition du ménage. Et donc l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. La composition du ménage est obtenu à partir de la base de données afférentes à la taxe d'habitation. Pour bénéficier du chèque énergie. Il faut donc avoir déclaré ses impôts et occuper un logement assujettis à la taxe d'habitation. Or l'imposition à la TH des résidents des Ehpads ne concerne que les EPHAD, à but non lucratif puisque les locaux des Ehpad à but lucratif sont d'imposer de leur côté à la cotisation foncière des entreprises, la CFE et s'agissant des Ehpads à but non lucratif seul sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation, les résidents ayant la disposition privative de leur logement au sein de l'Epad, c'est-à-dire sans restrictions importantes au droit de jouissance comme l'obligation de prendre leurs repas en commun ou encore le libre accès des chambres personnel actuellement seuls les résidents des Ehpad à but non lucratif ayant la disposition privative de leur logement reçoivent donc le chèque énergie actuellement. Les résidents des Ehpads à but non lucratif ayant la disposition privative de leur logement reçoivent un chèque énergie sous forme d'envoi automatique comme les autres ménages. Les résidents des autres structures eux sont également éligibles sous la forme d'une aide spécifique qu'érable via les questions léguées gestionnaire pardon auprès de l'Agence de services et de paiement. Enfin, dans le cas de la prochaine réforme du disque. Positif du chèque énergie en 2024 liée à la suppression de la taxe d'habitation, les modalités d'usage du chèque, notamment dans les structures présentant un rôle social d'accompagnement des personnes âgées pourrait être étudié. Je vous remercie. Merci madame la ministre et Madame Richer dispose encore de. D'une longue durée de réponse. Merci, monsieur le Président je bat un record presque Madame la Ministre je vous remercie pour ces précisions. Je tiens quand même à, à redire que les résidences seniors ont toute leur place. Elles sont une alternative comme les résidences autonomie entre le domicile et domicile et l'Epad, elles permettent de sécuriser les personnes qui font ce choix et de rompre l'isolement cet isolement reconnu comme néfaste pour nos aînés, et pour d'autres personnes. J'en tiens pour preuve puisque ma question émane aussi d'une résidence qui existe sur mon département et je je je veux mettre en avant cette résidence qui est porté par aussi Sylvie Olivier à Sancerre. Qui accueille 14 présidents issus de milieux différents qui répond au désir de résidence à taille humaine familiale puisqu'elle est complète, sans oublier que ces résidents sont créatrices d'emplois pérennes. Madame la Ministre puisque ces personnes perçoivent le chèque énergie, comment peut-on leur expliquer que l'option choisie n'est pas compatible avec le soutien du gouvernement. La liberté de choix que font les personnes accueillies la fraternité qu'elles y trouvent devrait nous conduire vous conduire à l'égalité de traitement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cher collègue, la parole est maintenant madame Michelle Gréaume pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. En 2008, le recensement a fait l'objet d'une réforme depuis cette date, il repose sur une collecte d'informations annuelle concernant successivement tous les territoires communaux ou d'une période de 5 ans. De cette comptabilisation de la population communale des cool le montant des financements accordés par l'État à chaque entité municipale. Or à l'usage ce système présente de nombreuses limites. D'abord le délai important avant la mise à jour de la population effectif des communes pénalise certaines collectivités qui ont vu leur population progresser ces dernières années mais ne bénéficient pas encore d'une revalorisation des dotations d'État des défaillances notables ont également été identifiées. Quant à la méthode du recensement qui biaise les résultats. Les agents recenseurs peuvent ne pas recevoir de réponse lorsqu'il se présente, il dépose alors un formulaire que les habitants doivent remplir sur le site du recensement dans un délai donné cela suppose que chacun ait accès à Internet puissent compléter les informations dans un délire restera alors que le site a déjà présenté plusieurs fois des pannes de plus, les consignes sont parfois perçue comme floue et par conséquent les informations renseignées erronée. Tous ces obstacles conduisent à un recensement souvent inférieurs à la réalité. La fiabilité du recensement reste donc aléatoires et cela a des conséquences non négligeables dans le versement des dotations financières aux communes. La réforme de 2008 avait prévu dans ces termes qu'il serait possible de faire évoluer le système dans le temps de procéder à une évaluation pour réajuster les modalités. Cette évaluation s'avère aujourd'hui nécessaire afin d'en déterminer les limites et d'ajuster son fonctionnement face à ces défaillances. Il faut répondre au mécontentement légitime des maires et des élus locaux, pour qui cet exercice peut être lourd de conséquences, madame la Ministre, comptez-vous procéder à une évaluation du recensement et quelle évolution envisagez-vous d'y apporter pour en améliorer la fiabilité merci. Madame la Ministre. Sur ce souvenir législatives de 2002 en réalité. Merci monsieur le président, madame la sénatrice, la méthode de recensement a été rénové en 2004 afin de réduire les délais de production des résultats par rapport à des recensement exhaustif entre lesquels il pouvait avoir un délai de 7 à 9 ans. De fournir des populations légales actualisée annuellement pour toutes les communes de France et de profiter des avancées méthodologiques pour réduire son coût pour les collectivités, mais aussi pour l'État. Les communes de moins de 10.000 habitants sont recensés exhaustivement une fois tous les 5 ans et toute la population est concernée. Leur population légale est actualisé tous les ans, avec les données de l'enquête de terrain et des données administratives. Les communes de plus de 10.000 habitants sont recensés tous les ans sur un échantillon de 8% des logements. La construction d'un nouveau lotissement ou d'un nouveau quartier et prise en compte dans l'actualisation des chiffres de population lorsqu'ils sont achevés sans attendre d'ailleurs la prochaine enquête sur le terrain les communes participent très activement à l'enquête de recensement et contribue aussi, de ce fait à l'élaboration des résultats, l'implication des communes sécurise le processus et garantit des résultats de qualité. Grâce à l'action de proximité des communes, le taux de réponse est extrêmement élevé, 95,2% en 2022. Pour toutes les communes de France, la population légale publié à la fin de l'année, reflète la situation effective. 3 ans auparavant. La population légale en vigueur au 1er janvier 2023 correspond à la situation du 1er janvier 2020. Ce décalage est un compromis nécessaires. Les méthodes de calcul des populations légales sont fondées sur l'obligation de garantir l'égalité de traitement de toutes les communes et ce décalage temporel entre. Date date d'entrée en vigueur et date de référence, permet de calculer une population à la même date pour toutes les communes. s'appuyant chaque année sur ces populations légales actualisée annuellement par l'Insee donc adapter depuis 2015, il est possible de répondre à l'enquête de recensement par Internet en 2022 70 % des personnes enquêter ont répondu d'ailleurs par Internet et le système informatique n'a connu que très peu d'incidents de très courte durée mais des discussions s'engageront à partir de mai 23, avec les associations d'élus pour justement parler des avantages et des inconvénients que pourraient avoir un calcul anticiper d'un an des populations légales par rapport à la situation actuelle à compter de même 2023. Je vous remercie. Madame la Ministre, je suis contente de savoir que, en mai 2023, il va y avoir des concertations concertant concernant sur recensement de la réforme de 2008, j'en suis heureuse je resterai vigilante par rapport à ça parce que sachez quand même que j'ai beaucoup d'élus locaux qui se plaignent du recensement aujourd'hui et du mode de fonctionnement informatique merci. Merci cher collègue. Maintenant, la parole est à Madame, Catherine Dumas pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance GPS est un groupement d'intérêt économique, constitué de 12 bailleurs sociaux il assure la surveillance de 165.000 logements et de plus de 500.000 habitants. Pour mener à bien ses activités. Ce groupement qui est d'ailleurs à but non lucratif dispose d'un budget annuel de de 18 millions d'euros qui est abondé par les bailleurs, membres du GIE et par une subvention de la Ville de Paris. Jusqu'au 1er janvier 2023, le GPS à bénéficier d'un rescrit obtenu en mai 2021 accordés par l'administration fiscale qui vise l'exonération de la TVA sur ces appels à cotisations. Il semblerait que la loi de finances initiale pour 2021 pourrait avoir modifié les dispositions légales sur lesquelles était fondée la demande de rescrit à compter du 1er janvier 2023, l'annulation de cette exonération risquerait d'entraîner une réduction des effectifs et des activités aussi afin de ne pas freiner son développement et d'assurer la sécurité des habitants des logements sociaux parisiens, je souhaiterais que l'exonération de TVA sur les appels à cotisations du GPS soit maintenu au travers d'un nouveau rescrit. dans ce cadre un dispositif transposer en droit interne dans le code général des impôts. Article 261 bé exonère de la TVA sous certaines conditions bien sûr les prestations de services effectués par les groupements autonomes de personnes au profit de leurs membres exerçant une activité exonérés ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA. La Cour de justice de l'Union européenne dans 2 arrêts de 2017 a précisé que s'agissant de la situation des membres exerçant des activités exonérés de la TVA, le dispositif ne peut s'appliquer qu'à la condition que les exonérations dont ils bénéficient relève uniquement de dispositifs d'exonération pour motif d'intérêt général prévues par la directive TVA. En revanche, l'exonération ne peut pas bénéficier à ceux des membres qui sont exonérés de la TVA sur d'autres fondements notamment, ce qui en sort les exonérations de la TVA dont bénéficient les activités financières et celle des bailleurs d'immeubles à la suite de ces arrêtés et dans un souci de sécurité juridique. La législation fiscale française a été mise en conformité avec la jurisprudence européenne et une nouvelle rédaction de l'article 261 B du code général des impôts est entrée en vigueur il y a quelques semaines le 1er janvier 2023. Désormais, seuls les services rendus par des groupements qui concourent directement et exclusivement. À la réalisation par leurs membres d'activités d'intérêt général exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de certaines dispositions de l'article 261 du code général des impôts peuvent être exonérés de la TVA. Ces activités ne comprennent pas l'allocation de logement qui est exonéré. Sur le fondement d'un autre dispositif, vous le savez le gypse j'ai soutient que c'est mon bailleurs sociaux restent éligibles à l'exonération prévu à l'article 261 B du code général des impôts ça demande fait encore l'objet aujourd'hui d'une instruction par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de rescrit couverts par le secret fiscal et il m'est donc très difficile d'aborder une situation fiscale individuelle dans le cadre d'une question orale mais ça vous le savez mieux que moi, madame la sénatrice Dumas.

le GPS a pu améliorer la situation sécuritaire. Sur Paris il contribue largement à la tranquillité résidentiel parmi d'ailleurs d'autres acteurs de la sécurité le gouvernement sur ce sujet d'intérêt général et sur ce cas particulier. Alors que nous entendent Mons cet après-midi l'examen en séance du projet de loi réformant notre système de retraite. J'attire justement votre attention sur la situation des retraités polypensionnés dont la carrière s'est partagé entre la France et la Suisse. Les ex-frontalier ayant effectué une partie de leur carrière en Suisse ont en effet la possibilité au moment de liquider leurs droits à la retraite de choisir de la de sauva de la percevoir Swat, sous la forme d'une rente, soit sous forme de capital. La question s'est longuement posé de l'assujettissement de ces retraits de suite suisse au paiement de la CSG CSG, de la CRDS et de la Casa. Pour les autorités fiscales françaises dès lors que le contribuable ex-frontalier était fiscalement domiciliée en France est affilié à un régime obligatoire de Sécurité sociale, celui-ci était redevable du versement de ces cotisations depuis le tribunal de Strasbourg. Suivant les conclusions de l'art et Nicolas de la CJCE à limiter le montant de ces prélèvements à hauteur du montant de la retraite française perçues par les retraités polypensionnés. Toutefois, d'après le code des impôts et de la lecture qu'en font les services fiscaux cette lecture ne s'appliquerait coûte retraité perçus sous des retraites perçues sous forme de rente et non à celle versée en capital d'après certaines associations de défense des droits des travailleurs frontaliers. Cette lecture pourrait être en contradiction avec la jurisprudence européenne et constituerait un frein à la libre circulation des travailleurs aussi, pourriez-vous nous indiquer comment le ministre. Entend-il lever cette ambiguïté et s'assurer que la pratique des services des services fiscaux français soit conforme au droit européen. Merci cher collègue. Et donc par l'État la Ministre délégué pour la réponse. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Schillinger vous m'interrogez au sujet des retraités polypensionnés qui réside en France mais qui ont effectué une partie de leur carrière en Suisse et qui touche à ce titre une pension française et une pension suisses. Le régime d'assujettissement se présente différemment selon que la pension suisses et versée en rente ou si elle fait l'objet au choix de la personne d'un versement en capital. Vous vous interrogez, à juste titre sur la cohérence de cette différence de traitement dans la première situation du versement rente de la pension suisses. La France s'est alignée sur la jurisprudence Nicolas. De la Cour de justice de l'Union européenne. Depuis un arrêt du Conseil d'État en date de 2019. Désormais, si la personne résident en France et qu'elles bénéficient de prestations maladie notamment versé par la sécurité sociale française. Alors la France peut définir l'assiette de contributions en prenant en compte la pension française et la pension suisses. Toutefois, en application de la jurisprudence de la Cour de justice. Le montant de ces contributions ne peut pas excéder le montant de la pension française. La sécurité sociale française ne peut effectivement pas précomptée des cotisations sur les rentes versées par l'institution de sécurité sociale suisse et c'est bien ce qu'applique l'administration fiscale dans la situation qui vous intéresse plus particulièrement du versement en capital de la pension suisses. La France ne suit pas la même procédure pour l'établissement des contributions sociales du le versement des pensions en capital et naturellement assujettis à la CSG comme celles qui sont versées en ronde d'ailleurs mais les modalités de fixation de la contribution ne peuvent pas être identique. On ne peut effectivement pas comparer une imposition assis sur une vedette en capital, qui fait l'objet d'un versement unique à une imposition qui correspond à une pension en rente versée chaque mois. Une application du plafonnement des cotisations. Montant de la rente mensuelle française aux pensions versées sous forme de capital ne serait pas fondées parce qu'elle reviendrait à une exonération de fait pour la rente versée C'est donc pour éviter justement cette situation qu'il est nécessaire d'assujettir les pensions versées sous forme de capital selon les modalités prévues par la législation française et indépendamment des principes issus de la jurisprudence européenne. Nicolas qui sont inapplicables à ce cas précis, je vous remercie. Merci madame la ministre et compliments pour votre capacité à résumer une question de cette complexité en 2 minutes 12. Madame Schillinger. C'est un dossier très technique. Je pense que je reviendrai souvent parce que c'est vrai que le, le dossier des frontaliers suisses et très très complexe et qu'il faudra vraiment une fois se pencher vraiment en profondeur. Merci madame la ministre. La suppression du service Info grève a été votée dans le cadre de la loi pacte du 22 mai 2019 relatives à la croissance et à la transformation des entreprises. Ce service devait être être remplacé par le guichet unique ah service aux grandes ambitions censé faciliter les démarches administratives des entreprises des autres entrepreneur des entrepreneurs, des experts comptables des avocats des notaires, des greffiers des tribunaux de commerce des organisations patronales des administrations publiques et enfin des collectivités territoriales. Opérationnel au 1er janvier 2002 2023 soit 3 ans après la promulgation de la loi est telle que cela a été annoncé. J'ai été saisi par les professionnels de la Moselle de l'incapacité de ce portail à traiter les demandes. Très complexe, suscitant des bug a répétition des données d'importance rejeté et des connexions hors délai. Le guichet n'a pas été au rendez-vous de ce qu'il était censé remplacer et cela dure toujours pour y pallier, la chambre des métiers de la Moselle a pris le relais mais à facturer des services qui aurait dû être gratuit les sommes ne sont pas négligeables, environ 200 euros par dossier. Un livre blanc des dysfonctionnements. Elle a même été rédigé par l'institut français des experts comptables et des commissaires aux comptes. C'est un préjudice considérable qui est affligé à notre économie qui concerne surtout les débutants, les repreneurs d'entreprises et leurs clients. Madame la Ministre, mes questions sont simples, pourquoi en sommes-nous arrivés là. Quelles solutions sont envisagées pour quelle date. Est-il prévu une plateforme performante juridiquement sécuritaire gratuites avec des remboursements légitime. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Herzog. Je n'aurai pas assez de deux minutes pour revenir sur l'histoire que j'assume évidemment des articles 1 et 2 de la loi pacte votée en mai 2019. À l'époque, j'ai pas assez de temps mais voilà je ne veux pas non plus qu'on refasse le match et l'histoire c'était pas si évident si centres de formalités de CFE. Un maquis incommensurable pour trouver son statut et et parvenir parfois entre des centaines de formulaires à ah on a créé son entreprise, donc il y avait bel et bien un besoin qu'il y ait des problématiques d'exécution. Je ne le nie pas, et j'ai à coeur de vous informer. Nous avons pris des mesures très ciblées, je rentre dans le vif du sujet pour améliorer les les travaux du guichet d'abord des travaux informatiques qui ont permis d'améliorer les délais de traitement des dossiers aujourd'hui un peu plus de 60% des créations sont ainsi traitées en moins d'une semaine et le stock de formalités de modifications mais aussi de cessation d'activité des premières semaines de janvier a été intégralement absorbé. Pour certaines formalités la voie papier qui constituaient la majorité des formalités a été temporairement temporairement en autorisé en complément de la voie dématérialisée de manière à offrir à l'usager, la voie la plus adaptée à ses besoins. Depuis le 20 février. Nous avons acté. L'ouverture d'une modalité supplémentaires pour réaliser les modifications et cessation. Avec notamment la mise en place le le retour d'un faux grève jusqu'au 30 juin prochain. Cette nouvelle voie d'accès pourrait concerner jusqu'à 15% du flux total des formalités. S'améliore le guichet unique a connu et je ne le nie pas quelques difficultés au démarrage, mais vu l'immensité de la tâche. Je peux nous pouvons comprendre ce qui est important c'est que ça s'améliore très rapidement après j'ai écouté attentivement votre question, je vais revenir sur la CMA je veux quand même vous dire que plus de 372.000 dossiers ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2023, dont plus de 200.000 créations dans un délai inférieur à une semaine concernant la CMA que vous mentionnez. Je suggère de prendre les coordonnées. Il n'a jamais été envisagé que malgré les difficultés, les entrepreneurs et à payer. Donc je suis à votre disposition et on s'en parle juste après. Enfin en tout cas je suis à votre disposition, parce que c'est pas normal je vous remercie. Entendu, chers collègues, vous avez quelques instants pour compléter. Bah, écoutez, je peux me satisfaire de cette réponse. C'est vrai que si les entreprises, c'est aussi l'économie. De notre pays et. C'est ça qu'il est urgent d'intervenir. On se, on se donne rendez vous tout à l'heure, merci. Entendu. La parole est maintenant à monsieur Jean-Claude en place. Merci monsieur le président. Madame la Ministre, chers collègues. Le gouvernement a annoncé que la rénovation énergétique des logements. Et l'éradication des passoires thermiques sont une priorité. Plusieurs dispositifs qui concourent comme celui de la prime rénovent. Toutefois, depuis sa création. Avec le projet de loi de finances 2020 le dispositif ma prévu rénovent rencontrent des difficultés. Le traitement des dossiers qu'on ait notamment des délais de traitement qui peuvent être long cas en cas d'erreurs techniques ou humaines lors de leur instruction. Si le gouvernement met en avant les chiffres positifs pour montrer la réussite de ce dispositif. Les difficultés ne sont pas marginales et ne permettent pas d'être aussi affirmatif. Elles engendrent des conséquences préjudiciables tant les entreprises d'artisanat du bâtiment, que des particuliers qui ont engagé des travaux de rénovation et particulièrement ceux aux revenus les plus modestes. Du fait des difficultés rencontrées par l'Anaes qui l'opérateur en charge de la gestion de l'eau et de la logistique de la distribution de ma prive rénovent les entreprises artisanales comme les particuliers sont en attente de paiement des aides prévues. Ils doivent donc supporter des avances de trésorerie dans un contexte économique difficile. Plus largement ces dysfonctionnements contribue à ralentir la rénovation énergétique du parc de logements et pénalise le secteur du bâtiment qui est déjà durement touchés par les conséquences de l'inflation sous les prix des matières premières. C'est pourquoi madame la ministre que j'ai plaisir à retrouver je vous demande quelles sont les solutions prévues par le gouvernement pour résorber ces délais d'instruction anormalement long et permettre ainsi l'accélération du versement des aides à la rénovation énergétique. Je vous remercie. que cette subvention principales aides de l'État pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique a permis de soutenir plus de 1,4 millions d'usagers depuis son lancement en janvier 2020 pour répondre à ces volumes très importants tout en traitant chaque demande individuelle pour s'assurer de son éligibilité Lana mobilise des équipes dédiées pour l'instruction et le paiement des dossiers autour d'une plateforme nationale dématérialisée dans un contexte de forte demande et de montée en puissance du dispositif avec l'extension des publics éligibles en 2021 et les primes exceptionnelles dans le cadre du plan de résilience gaz en 2022, certaines demandes ont pu rencontrer des difficultés à aboutir dans les délais habituels. Mais le nombre de cas est très limité. Si on le compare aux 630.000 primes engagé en 2022 par exemple l'se mobilisent fortement pour fluidifier le parcours usagers avec la mise en place d'une équipe dédiée aux situations les plus difficiles, les dossiers en difficulté font l'objet d'un suivi individualisé pour résoudre au plus vite les situations que vous décrivez la mais ainsi tous les moyens nécessaires en oeuvre. Pour s'assurer de la qualité de la rapidité du traitement des dossiers, le délai moyen de traitement observé pour un dossier MaPrimeRénov est inférieur à cinq semaines. Aujourd'hui, il ne s'agit donc pas de nier les difficultés encore une fois que vous soulignez, mais de les ramener à leurs justes proportions dans un dispositif dont le succès est indéniable et qui est un pilier de notre politique de rénovation énergétique. L'amélioration de l'information aux usagers est également une priorité avec l'objectif d'accompagner l'augmentation du volume de projets de rénovation la création du service public France rénove en 2022, complété par la montée en charge progressive de mon accompagnateur rénove en 2023 permettra de faciliter le parcours des ménages dans leur projet de rénovation entre autres initiatives pour répondre aux situations problématiques problématiques bien identifié l'Anna travaille avec la filière pour fluidifier le paiement des dossiers, je vous remercie. parce qu'il est important qu'ils se mettent en place les entreprises et les particuliers attendent. Je vous remercie. Merci cher collègue. Maintenant, la parole est à madame Hamel Gacquerre pour sa question. Monsieur le président, madame la ministre ma question porte sur l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques dans les années à venir et ses conséquences sur le secteur du logement. Réussir la transition écologique passe forcément par un plan en faveur de la lutte contre les passoires énergétiques, les dispositions de la loi climat et résilience vont dans ce sens en interdisant à la location les logements classés G, F d'ici 2025 et 2028. Concrètement, dès 2025, ce sont 600.000 logements classés G qui risque d'être retiré du marché locatif. Je suis favorable à l'instauration d'une obligation de rénovation et d'isolation, mais à certaines conditions. Le dispositif doit être juste et ne doit pas être punitif premières difficultés pour les propriétaires de biens classés F et j'ai l'ampleur et le coût des travaux dans un contexte où les matériaux et la main d'oeuvre viennent à manquer les dissuade donc d'engager des travaux. Ces mêmes propriétaires sont déjà confrontés à l'encadrement et au plafonnement des loyers, depuis l'été dernier à la hausse de la taxe foncière et aujourd'hui donc à cette obligation de rénovation énergétique la question de la capacité financière à réaliser des travaux se pose la puissance publique doit accompagner techniquement et financièrement. Or les moyens alloués aujourd'hui sont insuffisants et de nombreux propriétaires sont inéligibles au dispositif actuel. Autre effet de ces dispositions à laquelle nous sommes d'ores et déjà confrontée une explosion des ventes de logements F ou G et par conséquent un Net recul des logements loués. Près de 2 millions de logements risquent d'être retirés du menu du marché locatif dans les deux à venir à venir s'pardon. Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Ainsi la question également du calendrier se pose. du logement en France connaît déjà de nombreuses tensions avec une offre locative insuffisante et une demande en croissance. L'interdiction de mise en location des passoires énergétiques dans un délai court, risque d'aggraver les tensions sur le marché du locatif afin de garantir donc le droit au logement et d'éviter la crise du logement qui se dessine, je vous interpelle pour réviser l'échéancier de la loi afin de repousser l'interdiction de location des logements F à une date ultérieure et éventuellement envisager des dérogations en fonction de cas particuliers. Je vous demande également Madame la Ministre si des dispositions financières supplémentaires pour les propriétaires bailleurs sont envisagées afin de les aider, de les on les accompagner dans la rénovation énergétique de l'eau leur logement. Pardon, je vous remercie. progressive du niveau de performance énergétique minimal à atteindre dans le parc locatif social comme privés un seuil de 450 kWh par mètre carré et par an dès début 2023 la classe F en 2025, la Classe E E en 2028 et des en 2034 cette trajectoire découle de la loi climat et résilience de 2021. Elle constitue un élément indispensable à notre stratégie d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment avec un objectif de baisse des émissions de plus de 60%, à échéance 2023, qui découle de nos engagements européens. C'est une responsabilité réelle qui pèse sur les propriétaires de logements locatifs peu performant, environ 20% du parc locatif privé. Pour rappel, ce sont les locataires de ces passoires énergétiques qui sont aujourd'hui pénalisés, ils bénéficieront grâce aux travaux réalisés de plus de confort mais surtout d'une baisse de leurs charges d'énergie et c'est évidemment un point très important dans le contexte de prix élevés que nous connaissons actuellement les propriétaires bailleurs peuvent s'appuyer sur les dispositifs d'aides financières existantes qu'il s'agisse de MaPrimeRénov ou des certificats d'économie d'énergie pour mémoire l'ensemble des aides publiques et des CE. Pour la rénovation énergétique représente plaît près de 7 milliards d'euros en 2022. Un dispositif fiscal temporaire a également été introduit par la loi de finances rectificative pour 2022 et prévoit le doublement du plafond. Du déficit foncier en cas de travaux de rénovation énergétique pour accompagner les propriétaires bailleurs dans la rénovation de logements classés F ou G, le décret d'application doit être publié très prochainement en outre des évolutions substantielles visant à l'amélioration de l'accompagnement et du soutien aux propriétaires et aux propriétaires bailleurs ont été introduites grâce à la création du service public France rénovent les propriétaires-bailleurs ne manque d'après nous, donc pas d'outils pour respecter les échéances fixées. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Et maintenant, la parole est à monsieur Didier Marie pour sa question. Merci monsieur le président. Je souhaiterais Madame la Ministre appeler votre attention suite à une interpellation d'un certain nombre de maires de mon département qui connaissent des difficultés dans leur recherche d'un prestataire d'assurance pour couvrir leurs risques et dommages les prestataires d'assurance soit ne répondent pas aux appels d'offres soient propose des coûts très élevés que les communes comme celle du Petit-Quevilly en Seine-Maritime ne peuvent pas supporter, d'autant plus dans cette période d'inflation et d'explosion des coûts de l'énergie qui fragilise leur budget. À l'issue des procédures de marchés publics, certaines collectivités se retrouve donc dans l'incapacité de souscrire un contrat d'assurance, les laissant seuls face aux risques avec des conséquences éventuelles susceptible d'entraver le bon fonctionnement du service public local. Cette situation est le résultat d'une désaffection du marché des collectivités par les assureurs et fait peser un réel danger à moyen et long terme sur les collectivités. En effet, la multiplication des aléas climatiques notamment menace le Patrimoine des communes ne pourront pas porter seul. Les dépenses induites par ces éventuels événements. À titre d'exemple, certaines communes de mon département voient la moitié de leur superficie menacée par des risques d'inondations à l'horizon 2050, quand d'autres subissent le recul des falaises, ce sont des écoles, des médiathèques, des gymnases, des bâtiments municipaux nécessaires au bon fonctionnement des services publics de proximité que les collectivités doivent assurer pour garantir leur ouverture et la sécurité des agents qui travaillent ainsi que du public qui est accueilli. Bien que les collectivités locales tentent d'adapter leurs documents d'urbanisme et les constructions futures pour limiter les risques l'existant nécessite d'être protégée. Face à cette cette cette situation Madame la Ministre dans quelle mesure l'État. Par le biais d'un opérateur public ou d'une obligation de réponse aux marchés publics pour les compagnies d'assurance privées pourrait garantir la couverture assurantielle des collectivités locales à l'avenir, je vous remercie. Merci cher collègue là. Madame la ministre, votre réponse. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Marie, je partage votre préoccupation face aux difficultés rencontrées par certaines collectivités locales et intercommunalités pour souscrire une assurance de dommages aux biens en effet un nombre très réduit d'assureurs est aujourd'hui actif sur le marché de l'assurance des collectivités territoriales et doit répondre à près de 13.000 consultations publiques chaque année est le résultat de plusieurs facteurs cumulatifs l'existence de déséquilibre sur ce marché et le retrait d'assureurs, ces dernières années, en raison notamment de la hausse de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles. Face à cette situation, les services du ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont également engagé fin 2022 un cycle d'échange avec les principaux assureurs du marché de l'assurance des collectivités territoriales pour les alerter sur cette problématique des consultations approfondies des instances représentant les élus seront également menées parallèlement sous l'égide du président de la République. Le conseil de planification écologique et ce qui c'est les bases d'un important chantier de réflexion qui sera engagé cette année sur l'évolution du système assurantiel face à l'accroissement des effets liés au au dérèglement climatique. L'État a porté en 2021 à plus de 200 millions d'euros le budget alloué au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit le fonds Barnier qui peut être mobilisé par les collectivités pour financer des dépenses d'investissement afin de réaliser des études, des travaux ou des équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels. Il existe en effet une corrélation forte entre l'existence d'un plan de prévention du risque inondation sur un territoire et la fréquence des sinistres de la même manière que la mise en place d'un plan de prévention des inondations se traduit en moyenne par une réduction de 28% du coût des sinistres en tout état de cause la préoccupation que vous pointez est réel. Le gouvernement s'est saisi de cet enjeu important et nous ne manquerons pas de revenir vers vous, je vous remercie. Merci, madame la Ministre pour cette réponse. Il est heureux que le gouvernement les pris en considération cette difficulté. Ceci étant, au-delà de la concertation. Je pense qu'à un moment donné il faudra vraisemblablement amené de façon plus contraignantes les compagnies d'assurance à se préoccuper des situations des collectivités locales. Hein je vous remercie. Très bien. La parole maintenant monsieur Jean Marie misant pour sa question. Merci monsieur le président, madame la ministre, la dangerosité de notre parc d'autocars et as fait. L'accident depuis Seguin qui a fait date de notre pays car il a provoqué la mort de 43 personnes dans d'atroces conditions a effectivement mis en lumière, à défaut de conception de ces véhicules qui mériterait d'être corrigée dans les meilleurs délais afin, afin d'éviter d'autres pertes de vies humaines horriblement détruites. De fait aujourd'hui encore et après plusieurs drames le placement. Côte à côte du boîtier électrique et du réservoir à carburant tout à l'avant du car, dans une zone particulièrement exposée aux chocs en cas d'accident est tout simplement incompréhensible tant il est incontestablement hautement hautement meurtrier. En cas d'impact. L'explosion, qui se produit immanquablement aboutit en effet à un incendie et tandis que le véhicule s'embrase les passagers prisonnier de l'habitacle ne peuvent en réchapper et meurt brûlé vif. Par conséquent, allez-vous enfin tirer des enseignements de ces différents drames. Dont la cause est connue identifié et incontestable. Merci, cher collègue, la parole est à madame la Ministre délégué. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Mison en 2017. Le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre BE ATT a effectivement rendu un rapport d'enquête technique sur cet accident. La majorité des recommandations du BEAA ATT porte sur les modifications de règlements internationaux de la CE et de l'ONU concernant les véhicules en particulier les règlements traitant des caractéristiques de construction des autocars et des autobus et du comportement au feu de ces véhicules en 2017 et dès 2017 les autorités françaises ont demandé la création d'un groupe de travail international sur le comportement général des véhicules des autocars et autobus. En cas d'incendie ce groupe était présidé par la France. Il avait pour but d'établir un ou plusieurs projets de propositions de réglementation visant à rendre plus sur les véhicules en cas d'incendie. Les travaux du groupe ont abouti, ont permis que soit adopté et voté à l'ONU en 2021 puis en 2022 une série d'amendements au règlement concernés, il s'agira par exemple d'introduire de nouveaux tests sur l'inflammabilité des matériaux et d'améliorer les dispositifs de bris de vitres. Les premières dispositions entreront en vigueur sur les nouveaux types de véhicules à partir de septembre 2023. Je vous remercie. monsieur le président. Pas plus que vous mais la main Ministre je ne se de je ne souhaite à nouveau puis Ségur mais, hasard du calendrier ou pas, je viens d'apprendre que ce matin la cour d'appel de Bordeaux. Vient de. de. Rouvrir l'instruction de ce dossier. Justement. Concernant puis Seguin et parmi les raisons qu'elle évoque cette cour il y a notamment la conception du bus avec l'application du constructeur à savoir Mercedes. Je crois que, au-delà des accords il y a une question vitale

Merci, cher collègue, la parole maintenant Monsieur Henri Cabanel pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. La contamination de norovirus qui est à l'origine humaine et non animale est responsable de gastro-entérite hivernale après consommation de coquillages en janvier 2020, le gouvernement s'était engagé à améliorer le traitement des eaux usées en rappelant que les collectivités territoriales doivent maîtriser l'assainissement des eaux usées, que les contrôles concernant les rejets des stations d'épuration, les, les réseaux de plus d'eau pluviale pardon et les épandages dans des zones conchylicoles ferait partie des priorités adressée aux préfets et avait promis un retour d'expérience nationale permettant de définir les plans d'action de locaux. 17 zones de production ont été fermées en France cette année. Ces événements ont des conséquences majeures. Économiques pour de nombreuses entreprises le plus souvent familiales et de taille modeste. Le comité régional et au comité pardon national de la conchyliculture alerte sur l'urgence à agir. L'État doit manifester concrètement sa prise en considération de ces contaminations récurrente parfaitement identifiés et irrémédiable. Commun. Madame la ministre allez-vous concrétiser votre soutien à cette filière. Madame la ministre vous avez la parole. par un euro virus elle est due à plusieurs facteurs, une épidémie de gastro-entérite hivernale de fortes pluies qui ont entraîné un dysfonctionnement. Des systèmes d'assainissement et une forte augmentation de la population qui aggrave ses dysfonctionnements. Le gouvernement travaille donc sur la mise en conformité de ces systèmes d'assainissement. Mais ce sont tout simplement des chantiers le long et complexe face à l'urgence de la situation, nous travaillons avec les préfets sur 3 axes un lancer rapidement les travaux de renforcer leurs prescriptions lorsque les systèmes d'assainissement sont situés dans une zone dans une et puis troisièmement utiliser l'ensemble des mesures en matière de police de l'eau pour que les collectivités mettre rapidement aux normes les installations de collecte et de traitement des eaux usées, un état des lieux sera demandé pour lister les chantiers prioritaires et pour valoriser les bonnes pratiques ainsi que pour identifier les blocages, le gouvernement va également travailler sur un plan d'action avec les collectivités qui sera complémentaire à ces travaux. Un accompagnement financier pourrait être apportée aux conchyliculteurs via le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture ces aides à l'investissement pourront financer des bassins de mise à l'abri ou de purification des systèmes d'alerte des projets portés par les régions ou encore la constitution d'un système d'assurance pour laquelle l'État est prêt à accompagner la profession je vous remercie. Merci Madame la Ministre Monsieur Cabanel. Merci, madame la Ministre, de votre réponse. Vous savez comme moi que la dernière contamination a eu lieu en fin d'année entre Noël et jour de l'un ou chez moi en tout cas. Dans l'Hérault. Les conchyliculteurs font 60% de leur chiffre d'affaires. Et effectivement donc il y a. Une défiance des consommateurs qui a été entamée mais justement par rapport à à cette contamination et qui a. Un effet désastreux sur la reprise de la consommation de ces coquillages. Et vous l'avez signifié contrairement aux autres alias. Sanitaire. Il n'y a pas de dispositifs d'aide pour accompagner ce risque et la perte qui va bien sûr avec dans l'Hérault, les collectivités locales, que ce soit l'agglomération, que ça soit le département qui ça sur la région sont devenus un deux donc à la filière qui voit son avenir un petit peu. Sombre, donc j'espère que l'État aussi s'engagera à leur côtés je vous remercie. Comme bon nombre d'élus. J'ai été alertée il y a plusieurs semaines du projet de révision des normes de commercialisation européenne concernant les volailles de Chair. Comme vous ne l'ignorez pas, ce projet destructeur pour nos filières vise à changer les règles concernant l'étiquetage des modes d'élevage des volailles. Ces modifications ont un objectif clair et scélérat, à savoir organiser l'opacité en entretenant le flou sur les modes d'élevage de manière à ce que le consommateur ne soit plus en capacité d'identifier clairement l'origine et le mode d'élevage du produit qu'il a dans son assiette. Ce manque de transparence et de traçabilité joue au détriment de pays vertueux, comme la France et permet à d'autres pays n'ayant pour seul horizon que le rendement de ne pas avoir à rendre de comptes sur leur mode d'élevage. Tout comme l'ensemble de la filière. Je tiens à exprimer ma profonde opposition à ce projet. Je rappelle que les normes actuelles. Établissent une segmentation et un étiquetage clair en ce qu'elle permette aux productions de volailles. Alternatives d'être mieux connus des consommateurs et trouver une place sur le marché. Vous le savez madame la Ministre, la France est le pays européen avec la plus grande production de volailles alternative. Et le département de la Sarthe participe pleinement à ce rayonnement de fait, cet étiquetage est particulièrement important en Sarthe que je représente ou les productions fermières élevées. En liberté ont une place importante puisqu'elle représente à elle seule, au moins 20% de la production française, notamment via les productions AOC, Label rouge et bio. Madame la ministre, pouvez vous rendre compte. À ce stade à la représentation nationale des actions menées par le gouvernement auprès de la Commission européenne afin de garantir à nos producteurs que l'étiquetage actuellement en vigueur. Puisse perdurer. Merci cher collègue. Madame le Ministre votre réponse s'il vous plaît. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Cozic une réforme a été initié par la Commission européenne dans le courant de l'année 2022 et le projet de texte transmis en janvier aux États, a suscité de fortes inquiétudes de la part des professionnels sur 2 points l'obligation d'étiqueter toute viande de canard ou d'oie issu de la production de foie gras avec la mention issus de foie gras et deuxièmement une dérégulation de l'usage des mentions valorisantes pour l'étiquetage de la viande de volaille jusqu'alors limitée à une liste fermée de 5 mentions valorisantes. Ce qui aurait eu pour effet de décupler les risques de concurrence déloyale entre opérateurs et de tromperie des consommateurs, il faut souligner que ces normes revêtent un intérêt économique majeur pour la filière volailles. elles ont permis depuis leur instauration d'offrir une meilleure visibilité aux productions de volailles extensive en plein air par rapport aux autres pays européens la filière volaille française se caractérise ainsi par une forte segmentation du marché plein air notamment en signe de qualité et de Label rouge, nous avons supporté les bons messages et ce travail porte ses fruits aujourd'hui puisque la Commission européenne vient de soumettre à l'avis des États membres. Un projet de texte qui prend en compte les demandes de la France est satisfait les professionnels avec le retrait de l'obligation d'étiquetage des viandes avec la mention issus de foie gras et une rédaction de compromis qui protège et maintient l'exclusivité de l'utilisation des mentions plein air. Il convient toutefois de rester prudent dans la mesure où ce projet de texte doit encore passer plusieurs étapes avant sa publication dans quelques semaines, le travail se poursuit donc désormais pour consolider le résultat positif qui se profile. Je vous remercie. Merci madame la ministre, chers collègues. Il vous reste quelques instants mais pas indispensable madame Loyer. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, madame Amice, mes chers collègues Madame Miss ma question porte en fait sur les montants des indemnisations forfaitaires des bovins ayant fait l'objet d'un abattage pour diagnostic sanitaire ces abattages sont encadrées par un arrêté de juin 2009 qui fixe les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose la tuberculose bovine ou caprine. Les acteurs de la filière ont sollicité, monsieur le ministre de l'Agriculture depuis plusieurs mois leur requête se fonde notamment sur l'évolution des prix actuels et sur l'indexation des fameux coup de coûts de production dans le cadre de la loi Egalim. Cette demande vise en fait à majorer l'indemnisation entre 2000 et 2500 euros par bovin pour plus de de plus de 24 mois non inscrit au Livre généalogique. la situation serait bloqué Madame la Ministre par la direction du budget qui aurait mis en avant le coup d'une autre crise sanitaire, la grippe aviaire qui auraient consommé l'ensemble des enveloppes budgétaires, y compris celle réservée donc au paiement des abattages pour diagnostic reportant ces valorisations pour la campagne de prophylaxie, 2023 2024. En outre, aucune rétroactivité ne serait envisagée pour les éleveurs ayant fait déjà abattus, des bovins sur la campagne de prophylaxie actuel si tel est le cas, cela porterait un réel coup de frein à l'action sanitaire majeur à la fois des directions départementales de la populaire. Protection des populations, les groupements de défense sanitaire. Les vétérinaires et tous leurs partenaires qui sont engagés depuis de longs mois, notamment pour éradiquer la et nous le savons tous retard pris dans la gestion des abattages génère une hausse du nombre des foyers contaminant et diminue d'autant. L'efficacité du dispositif. Pourriez-vous donc nous préciser Madame la Ministre parce qu'il me semble qu'il y a eu des dispositions récentes les. Les efforts que pourrait faire le gouvernement, le gouvernement pour permettre une revalorisation de ces indemnisations des bovins abattus rapidement et, et notamment une revalorisation à hauteur des montants évoqués et avec et, avec ce principe de rétroactivité au 1er janvier de l'année. Je vous remercie, madame la Ministre. Merci cher collègue. Et donc la ministre que répondre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Loisier. La tuberculose bovine peut contaminer tous les mammifères, dont l'homme l'assainissement des troupeaux est donc indispensable pour éviter la diffusion de la maladie et ainsi protéger les élevages français, et donc la santé publique. Il faut rappeler l'importance des actions de biosécurité qui permettent de réduire drastiquement le risque de contamination entre entre exploitation ou par la faune sauvage, une formation à la biosécurité est dorénavant obligatoire pour le recouvrement de la qualification indemne d'un troupeau ayant été comptabilité et l'État a mobilisé 3,5 millions d'euros dans le cadre de France relance pour les financer. Par ailleurs, 2 points. Premièrement, les talents sont 2023 une expérimentation sur la faisabilité de la vaccination des blaireaux comme en Irlande et deuxièmement l'autorisation du recours du test en prise de sang, réduit la durée de blocage des exploitations et réduit le nombre d'abattages diagnostic diagnostic d'animaux déclarés suspects. Grâce à une analyse de risques. Seules les exploitations de 20 départements sont dorénavant soumis à une surveillance renforcée. Il n'existe plus de surveillance minimale sur tout le territoire français. J'en viens au point spécifique de votre question sur lequel Marc Fesneau a eu l'occasion d'apporter des précisions lors du et a un niveau d'indemnisation trop faible des abattages diagnostiquée. Nuit véritablement à la qualité de la surveillance dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, des animaux abattus dans le cadre d'abattage diagnostic sont indemnisés sur la base de forfait avec l'évolution des cours de la viande et des cours de production les forfaits fixée par l'arrêté en vigueur nécessité une mise mise à jour de plus, au regard des risques de sous-déclaration qui résulte du décalage entre la valeur réelle et le montant. Des animaux. Un nouvel arrêté cosigné par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire vient de revaloriser les forfaits de 100 euros à 600 euros en fonction des catégories d'animaux. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Et donc nous passons à la question de madame les guide, ce qui a la parole. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais aller. Attirer votre attention sur une situation préoccupante. L'inefficacité en droit et en fait du régime juridique de sanction des infractions commises par les poids lourds circulant sur des voies interdite aux véhicules lourds. Force est de constater qu'en dépit de la loi du 24 septembre 2019 d'orientation des mobilités qui autorise l'installation de radars poids lourds pour faciliter la constatation et la verbalisation de ces infractions nos communes demeure à ce jour largement impuissante pour faire respecter les arrêtés municipaux régulant la circulation des poids lourds. Et si dans une réponse au Sénat du 2 février 2022. Le gouvernement évoqué la possibilité prochaine d'une installation de radars poids lourds fixe à l'initiative des maires. Je ne peux que déplorer que faute de clarification législative et réglementaire dédié l'état actuel du droit ne permet toujours pas la verbalisation effective de ces derniers en effet la différence des dispositions législatives en matière de vidéo-verbalisation des nuisances sonores excessives sur la route introduite par cette même loi de décembre 2019, les radars poids lourds n'ont toujours pas fait l'objet d'une expérimentation en lien avec les collectivités. De même la circulation de poids lourds sur des voies qui leur sont interdites, ne figure toujours pas à la liste des infractions vidéo verbalisable énumérés à l'article R. 130 11 du code de la route. Les élus locaux peuvent librement faire des arrêtés municipaux interdisant l'accès de ses poids lourds à certaines voix sensible mais le reste et finalement dépourvue de moyens efficaces pour les faire respecter. Je souhaiterais savoir comment vous envisagez de procéder aux clarifications législatives et réglementaires requises et d'autoriser dans les meilleurs délais au moins à titre expérimental la vidéo-verbalisation du trafic des poids lourds dans les collectivités locales de nombreuses communes sont prêtes à prendre part à une telle expérimentation, je vous remercie de votre attention. Madame la ministre. Votre réponse à cette intéressante question. Si monsieur le Président Madame la sénatrice guider ce gouvernement est particulièrement attaché et de la circulation, la police de circulation, de moyens juridiques et techniques pour faire respecter efficacement les règles de la sécurité routière dans leur agglomération comme vous le rappelez, cela s'est traduit dans la loi d'orientation des mobilités par la compétence attribuée aux maires, de décider de l'installation de radars pour le contrôle du respect des voies réservées du tonnage des poids lourds et des zones à faibles émissions. Les délais nécessaires à la définition et au développement technique d'équipements radar fiable dédiés au contrôle des voies réservées des ZFE et des poids lourds. La seule option disponible à court terme pour mettre en oeuvre un contrôle sans interception alliant efficacité de la répression et facilité de mise en place repose sur la vidéo-verbalisation elle autorise normalement les policiers municipaux et les gardes champêtres à constater les infractions sans interception après visionnage en Direct des images issues d'un système de vidéo-, protection des modifications réglementaires sont d'ores et déjà engagés par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer afin d'étendre le périmètre des infractions constatable sans interception listé à l'article L 121 tiré 6 du code de la route aux interdictions et restrictions de circulation prévues par la réglementation sur le poids des véhicules mais aussi pour élargir l'accès au système d'immatriculation des véhicules des policiers municipaux afin qu'ils puissent obtenir les données relatives à la catégorie des véhicules. La publication de ces textes permettra de finaliser le cadre juridique mais ne permettra malheureusement pas de mettre en place immédiatement les appareils de contrôle en effet ces appareils ont pour finalité d'identifier de verbaliser des usagers de la route en infraction, ils doivent donc disposer de toutes les sécurités de toutes les homologations nécessaires pour que ce nouveau système ne comporte pas de faille, les appareils devront notamment être connecté à l'Agence nationale de traitement automatisé des 1 francs des infractions je peux vous indiquer que la certification des équipements pilotée par mon collègue en charge des Transports Clément Beaune est prévue pour mi-2023. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous savez que la seule modalité de verbalisation des poids lourds en infraction demeure à ce jour l'interception de véhicules pris sur le fait par des services de police et de gendarmerie déjà très. Très sollicités Très sollicités par ailleurs ce cap non normatif est ainsi très restrictif et peu adapté aux réalités pratiques pour être efficace aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Bruillet, c'est à vous pour votre question. Merci monsieur le président, madame la ministre je souhaite vous interroger sur la notion de trouble grave à leur public dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat d'engagement républicain. Le premier engagement du contrat d'engagement républicain précise le respect des lois de la République s'imposent aux associations et fondations qui ne doivent entreprendre ni incité à aucune action manifestement contraire à la loi violente ou susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public présentant cette loi à l'Assemblée nationale, le 1er février 21. Le ministre de l'Intérieur déclarait ce texte combat surtout et avant tout les idéologies singulièrement l'idéologie islamiste, même si elle n'est pas la seule. Il ajoutait grâce au contrat d'engagement, l'État et les collectivités auront à leur main un outil juridique le Haut Conseil à la vie associative dans ces dernières. Avis a estimé que le contrat d'engagement républicain tendait à confier à l'administration un pouvoir d'interprétation et de sanctions très large sans information claire préalable et est obligatoire sur les voies de recours susceptible d'être exercée par les associations et fondations. Madame la ministre, en septembre 2022, le préfet de la Vienne. Jean-Marie Girier sommé la ville de Poitiers. La communauté urbaine de retirer leurs subventions au village des alternatives organisée par l'association Alternatiba Poitiers. D'après le journal Libération, cette décision aurait été prise par le préfet en raison d'une formation consacrée à la désobéissance civile qui serait manifestement incompatible avec le contrat d'engagement républicain je souhaite savoir si la formation à la désobéissance civile est constitutif de troubles graves à l'ordre public. Si oui, pouvez-vous préciser sur quelle définition de troubles graves leur public. Le préfet de la Vienne se fonde pour une telle décision. Enfin, je souhaite que vous m'indiquer si la dénonciation non-violente de l'inaction ou de l'insuffisance d'action écologique est une idéologie à combattre au même titre que l'idéologie islamiste. Merci, cher collègue, la parole est à madame la ministre. par la souscription du contrat d'engagement républicain C E R à respecter un ensemble de principes républicains annexée au décret d'application du 31 décembre 2021. Le 1er de ses engagements impose aux associations de d'entreprendre ni d'inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public si une association ne respecte pas ses engagements. L'autorité administrative qui lui a attribué une subvention doit procéder à son retrait après une procédure contradictoire. Une subvention a été accordée par le conseil municipal de Poitiers à l'association Alternatiba Poitiers afin d'organiser un village des alternatives, alors même qu'il est très prévu que des ateliers de désobéissance civile et lieu dans ce cadre. Le préfet de la Vienne informé la maire de Poitiers, qui était nécessaire, que le conseil municipal engage la procédure de retrait de la subvention car de tels ateliers serait manifestement incompatible avec le 1er engagement du CER. Le conseil municipal a pris une nouvelle délibération, refusant d'engager la procédure de retrait dès lors en application des dispositions de l'article L 21 31 tirer 6 du code général des collectivités territoriales le préfet a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision, l'injonction faite par le préfet de retirer la subvention versée à cette association ne reposait pas sur le motif que les formations à la désobéissance civile constitue par principe des troubles graves à l'ordre public. Mais sur le motif que ces activités peuvent constituer une incitation à des à des actions manifestement contraire à la loi. Il convient de rappeler que même avant l'entrée en vigueur du CER la jurisprudence du Conseil d'État estimé que de telles actions justifier le retrait du financement public accordé aux associations concernées ainsi la démarche du préfet de la Vienne ne fait que traduire l'application de la volonté du législateur qui par l'instauration de ce C. E R a entendu empêcher que l'argent public serve à ce qu'une association incite à des actions manifestement contraire à la loi. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Monsieur, Monsieur Boyer, vous ne vous reste deux ou trois secondes. Merci, monsieur le Président, juste pour dire que c'est un comble, qu'une loi pour lutter contre l'idéologie islamiste serve à affecter une des plus grandes lois de liberté de notre pays. La loi 1901. Madame Boyer, c'est à vous. Si Monsieur le Président Madame la Ministre alors que vous avez toujours crié au scandale lorsqu'il était fait un lien entre immigration et délinquance. Le ministre de l'Intérieur a reconnu l'été dernier et je le cite, qu'il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. 48% des gens interpellés pour des actes de telles hein quand ça Paris 55 à Marseille, 39 à Lyon sont des étrangers. Comment ne pas évoquer le meurtre qui a ému toute la France, celui de la petite Lola sauvagement agressé par une ressortissante algérienne qui n'aurait pas dû être sur le sol français. À défaut de position d'un type de séjour elle avait fait l'objet d'une OQTF, vous y voyez des faits divers. J'y vois des faits de société ces OQTF ne sont pas respectées sur le 1er trimestre de l'année 2021, seuls 56. 5. 6 % d'entre elles ont ont été exécutés et encore on ne sait pas où ces personnes. Ont fait l'objet de ce retour chez elle, selon les chiffres du parquet de Paris, il estime que 75% des mineurs jugés sont encore des mineurs étrangers. Dans un contexte de surpopulation carcérale avec des étrangers qui représentent 24% de la population carcérale en 2020 alors qu'ils ne sont que 7, 4% en France. Ce, ce problème est vraiment important, c'est pourquoi je souhaite de nouveau obtenir davantage d'informations sur le nombre d'étrangers condamnés le nom d'étrangers incarcérés leur nationalité. Le nombre d'expulsions réellement exécutées ainsi que la liste de leurs crimes et délits concernant également ces crimes, notamment sur les attaques à l'arme blanche je demande une cartographie détaillée et précise, j'indique que les victimes d'agression à l'arme branches sont montés à 44.000 entre 2015 et 2017, soit plus de 120 victimes par jour en moyenne, selon les chiffres que vous avez vous-même communiqué. J'y ajoute aussi que je souhaite obtenir le profil des auteurs et les victimes afin de pouvoir établir un plan d'action et d'éviter que ces attaques se poursuivaient se multiplient. La représentation nationale doit connaître précisément quelle est la cartographie de cette violence pour en tirer tous les enseignements, merci. Merci cher collègue. Madame la Ministre c'est ça. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Boyer. Comme vous l'avez indiqué l'éloignement des étrangers. Une menace pour l'ordre public, constitue une priorité constante de l'action des services de l'État des protocoles entre les établissements pénitentiaires et les préfectures ont été signés afin de faciliter l'identification de l'étranger avant la fin de son incarcération et son éloignement. Dès la levée d'écrou par un partage d'informations entre ces autorités 2 opérations se sont succédé au second semestre 2021 et au 1er semestre 2022, ciblant notamment les étrangers en situation irrégulière sortant de prison. Elles ont permis d'éloigner de 1815 étrangers en situation irrégulière et dont le profil évoquait des risques de troubles à l'ordre public depuis le 18 octobre 2020, c'est 317 étrangers inscrits au FSPRT radicalisé au constituant une menace grave lors de public qui ont été éloignées par une instruction du 3 août 2022. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rappelé aux préfets la nécessité de placer prioritairement en rétention administrative. Les étrangers inscrits au FSPRT ou dont le profil évoque des risques de troubles à l'ordre public, 88% des trajets en centre de rétention administrative répondent à ce profil et se trouve donc en en instance d'éloignement pour renforcer les capacités mobilisées au service de cette action. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a accepté d'amender la trajectoire budgétaire inscrite dans la Lopmi à hauteur de 60 millions d'euros par an pour développer des capacités de rétention et est porter à un niveau jamais atteint. S'agissant des attaques à l'arme blanche statistique institutionnel du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Le SS M. S. il ne recense pas ce type de phénomène en effet la qualification des infractions issu du code pénal ne permet pas de faire cette distinction et dans la classification historique des infractions établies établies par le ministère de l'Intérieur, elle n'est faite que dans le cadre de vols violents. S'agissant de la part des étrangers dans la délinquance. Les éléments statistiques du SPS M. S. ils font apparaître la part des étrangers non par pays mais par grandes régions d'origine le Maghreb, l'UE l'Asie et cetera dans les personnes mises en cause, comme dans les victimes, je vous remercie. suivi. Concernant les autres chiffre ce que vous citez, on les a déjà mais je vous ai demander de plus précis, c'est de ça dont nous avons besoin pour travailler. Madame, je vous remercie. Très bien je vais suspendre la séance. Elle va être reprise à 14h 30 pour l'examen du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, la séance est suspendue.